Si cette mesure est de bon sens, elle n’a toutefois pas été assortie d’une recommandation de propreté pour les jeunes enfants entrant en maternelle. Or de nombreux maires m’ont fait part de l’absence de plus en plus fréquente de propreté de cette classe d’âge, certains enfants arrivant même avec des couches.

Dans l’article 2 du décret n° 2018-152 du 1 mars 2018, il est indiqué que « les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l’assistance au personnel enseignant pour l’accueil et l’hygiène des enfants des classes maternelles ou enfantines, ainsi que de la préparation et la mise en état de la propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants ». Comme, il est indiqué dans cet article, ces agents sont chargés d’apporter assistance pour l’hygiène des enfants. En aucun cas, cela ne signifie que leur rôle est d’apprendre aux élèves à devenir propres. Les communes investissent massivement pour faire monter en compétences leurs Atsem et revaloriser le travail essentiel qu’elles ou ils effectuent au quotidien auprès de nos enfants. Ces agents territoriaux ont obtenu en 2018 une amélioration dans le déroulement de leur carrière, mais là, madame la secrétaire d’État, leur moral est au plus bas. Il n’est en aucun cas question pour elles et pour eux de ne plus prendre soin de l’hygiène de nos enfants, mais leurs journées ne peuvent

Ils sont en général scolarisés la journée entière. Je dis bien « en général », et je m’en explique. L’école maternelle prend bien évidemment en compte les besoins physiologiques et de développement de chaque enfant. Elle participe à son éducation à l’hygiène en lien avec les familles

tenir compte du jeune âge des enfants, le législateur a prévu la possibilité pour les responsables légaux de solliciter une dérogation à l’obligation d’assiduité pour les enfants scolarisés en classe de petite section se traduisant par un aménagement des horaires, notamment l’après-midi.

Une institutrice souhaitant devenir directrice d’école élémentaire doit s’inscrire sur une liste départementale d’aptitude aux fonctions de directeur d’école. L’ancienneté requise de services effectifs est de deux ans et les candidatures parviennent à l’inspection académique revêtues de l’avis motivé de l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription. Une commission d’entretien, composée de l’inspecteur d’académie ou de son représentant, d’un inspecteur et d’un directeur d’école, émet un avis après étude du dossier et entretien avec le candidat. L’inspection académique arrête alors la liste d’aptitude après avis de la commission administrative paritaire départementale. Il s’agit d’une procédure nationale extrêmement codifiée,

notamment en ce qui concerne les ressources humaines. En effet, dans la ruralité, les élus locaux travaillent en lien très étroit et constant avec les directeurs d’école, dans le souci de maintenir dans leur commune la qualité du service public de l’éducation. D’ailleurs, le Président de la République avait bien compris le rôle essentiel du maire en prenant l’engagement, dès 2019, qu’aucune fermeture de classe ne pourrait se faire sans l’accord préalable de ce dernier. Dans le cadre du plan ruralité, lancé par la Première ministre le 31 mars 2023, l’un des axes de travail pourrait être, en accord avec les préconisations de l’inspection générale, l’amélioration de la politique de recrutement des directeurs d’école.

accord avec l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription, en remplacement de la directrice titulaire absente pour congé de maternité prolongé. Cette institutrice a su assurer une continuité administrative, pédagogique et relationnelle

territoires ruraux. Dans cette perspective, le 31 mars dernier, la Première ministre et le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse ont annoncé l’élargissement de la démarche des Territoires éducatifs ruraux à l’ensemble des départements ruraux. Cette extension s’inscrit dans un plan ruralité beaucoup plus large qui vise à garantir l’amélioration durable de la qualité du service public de l’éducation au sein de ces territoires. La loi du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice ou de directeur d’école prévoit que le directeur d’école est nommé parmi les personnes inscrites sur une liste d’aptitude. Ne peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude que les instituteurs et professeurs des écoles qui justifient de trois années d’enseignement ou d’une année au moins d’exercice de la fonction de directeur d’école, et ont suivi une formation à la fonction de directeur d’école. Dans le cadre de vacance d’emplois de directeur d’école, des instituteurs et des professeurs des écoles non inscrits sur la liste d’aptitude peuvent aussi être nommés à leur demande, dans des conditions définies par décret. Un décret publié cet été précise les modalités de recrutement des directeurs d’école : une liste d’aptitude à l’emploi de directeur d’école est établie chaque année dans chaque département par le directeur académique des services de l’éducation nationale. Une commission départementale formule ses avis sur les candidatures, après examen des dossiers et un entretien avec chaque candidat. Les mutations et affectations des directeurs d’école peuvent s’effectuer, selon le mouvement national et intradépartemental, sur l’ensemble des postes de direction déclarés vacants pour une rentrée scolaire, ainsi que sur postes à profil aux niveaux national, d’une part, et intradépartemental, d’autre part. Dans ce cadre sont proposés aux enseignants des postes qui requièrent des compétences particulières, en lien avec le projet de l’école. La parole est à M. Max Brisson,

motif qui ne tient pas compte du manque de reconnaissance par le ministère de nombreuses associations où la pratique est intensive ; l’itinérance ou l’éloignement, motif qui n’intègre pas le caractère imprévisible des mobilités, contraintes dans une fenêtre de dépôt entre le 1 mars et le 31 mai. et le 31 mai. Si ces trois premiers motifs, par leurs restrictions, soulignent votre volonté de « scolarisation à tout prix », c’est bien le quatrième motif qui justifie ma question : « Une situation propre à l’enfant motivant un projet éducatif. » Ce motif laisse

délivrée par les services académiques, pour des motifs tirés de la situation de l’enfant et limitativement définis par la loi. Au titre de l’année scolaire 2023-2024, un peu plus de 50 000 demandes d’autorisation d’IEF ont été instruites. Elles ont donné lieu à une large majorité d’autorisations 89 %, soit 43 907 autorisations –, essentiellement des autorisations de plein droit, pour 72 % d’entre elles, et 28 % au titre de l’un des quatre motifs prévus par la loi. Ces demandes ont donc donné lieu à une minorité de refus.

Il est à noter que le Conseil d’État a clarifié dans plusieurs décisions du 13 décembre 2022 les conditions d’application de la loi. Lorsqu’ils sont saisis d’une demande d’autorisation d’IEF fondée sur l’un des quatre motifs d’autorisation définis par la loi, les services académiques doivent rechercher, au vu de la situation de l’enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction dans un établissement scolaire, d’une part, et de son instruction dans la famille selon les modalités exposées par la demande, d’autre part. À l’issue de cet examen, Ainsi, il ne s’agit pas d’interdire sans discernement tous les dispositifs d’instruction en famille et de porter atteinte aux pratiques positives. À cet égard, les services du ministère de l’éducation nationale accompagnent les services académiques dans la mise en œuvre du nouveau régime d’autorisation d’instruction en famille.

avec des annonces que je salue sur l’abaya ou encore sur le harcèlement scolaire, véritables fléaux pour notre école républicaine. Cependant, après le temps de la communication vient celui du bilan de la rentrée. Des dysfonctionnements et un manque criant de moyens sont encore à souligner, comme au collège René-Cassin, à Tourrette-Levens, dans le département des Alpes-Maritimes. Cet établissement souffre d’un sous-effectif chronique, comme ont pu le souligner, auprès de la rectrice d’académie, les maires concernés d’Aspremont, de Colomars, de Saint-Blaise, de Tourrette-Levens, de Duranus et de Levens, ou encore les députés Éric Ciotti et Christelle D’Intorni. conseillers principaux d’éducation (CPE) adjoints : autant de lacunes portées à la connaissance de l’administration, qui n’a pourtant donné aucune suite. Il aura fallu une grève de ce collège et des opérations « coup de poing » pour que vous preniez enfin, semble-t-il, quelques décisions. Le rectorat a ainsi annoncé voilà quelques jours du personnel supplémentaire à la rentrée de 2024. Madame la secrétaire d’État, réparer l’école, c’est non pas répondre à l’urgence, mais remanier de manière pérenne. l’enquête singulière réalisée par le syndicat Unsa, qui est loin d’être le plus radical, le prouve : l’académie de Nice est en souffrance. Aussi, pouvez-vous confirmer les créations de postes annoncées ? Allez-vous redonner aux Alpes-Maritimes, mais aussi à l’ensemble du pays, les moyens nécessaires à

d’actualité au Gouvernement. Plus précisément, la situation du collège René-Cassin fait l’objet d’un suivi particulièrement attentif de la part du rectorat de l’académie de Nice depuis plusieurs années. L’accroissement important du nombre d’élèves au cours des dernières années a conduit à des extensions de bâtiments pour permettre l’accueil des élèves en classe dans les meilleures conditions et renforcer les conditions d’encadrement. À l’issue d’audiences organisées au mois de juillet, puis au début du mois de septembre 2023, des moyens supplémentaires ont été accordés, avec la création d’une division supplémentaire et d’un

avec effet immédiat, le recrutement supplémentaire d’un assistant d’éducation et d’un personnel administratif ; à compter de la rentrée scolaire 2024, la création d’un second emploi de CPE ; la stricte limitation des dérogations à l’affectation au collège aux seules demandes de droit. suite au dialogue engagé, la rectrice a renouvelé sa confiance dans toute la communauté éducative, ce qui a permis à l’établissement de fonctionner de nouveau de manière apaisée. Il convient d’ajouter que le conseil départemental des Alpes-Maritimes a donné son accord à la construction d’un nouveau collège, qui devrait ouvrir ses portes à la rentrée scolaire de 2026. Monsieur le sénateur, je vous assure que le rectorat demeure tout particulièrement vigilant sur la situation du collège René-Cassin

et de la formation professionnels. Madame la secrétaire d’État, je souhaite attirer votre attention sur les conséquences de la baisse du niveau de prise en charge des contrats d’apprentissage récemment annoncée par le Gouvernement par l’intermédiaire de son opérateur France Compétences. Après un premier rabais de 2,7 % opéré en septembre 2022, un nouveau tour de vis, de 5 % cette fois-ci, va venir encore diminuer le financement des quelque 850 000 contrats signés chaque année par des jeunes. Cette décision est regrettable, tant le modèle de l’apprentissage a prouvé son attractivité et ses effets auprès de milliers de jeunes âgés de 16 ans à 29 ans. Les efforts consentis par le Gouvernement depuis 2018 leur ont ainsi permis de bénéficier de solutions pertinentes pour leur formation et leur insertion professionnelle auprès des 137 centres de formation d’apprentis (CFA) répartis sur tout le territoire. La baisse annoncée va inévitablement dégrader l’accessibilité de ces formations sur le plan financier. Le coût des contrats est appelé à connaître une hausse de 10 % en moyenne : ainsi, un CAP en boulangerie verra son niveau de prise en charge passer de 6 683 euros à 6 015 euros. De nombreuses autres formations professionnalisantes devraient par ailleurs devenir rapidement déficitaires, encourageant ainsi les CFA à les supprimer de leur catalogue de formation, et ce même si nombre d’entre elles permettent de pourvoir des métiers en tension. Métallurgistes, couvreurs-zingueurs, carreleurs, carrossiers : la liste est longue ! Par cette décision, l’État semble se désengager de son action en faveur de l’insertion des publics les plus éloignés de l’emploi. Il s’éloigne des objectifs de la politique d’apprentissage qu’il s’était fixés, et prend le risque de créer un choc sur l’offre et la qualité des formations. Nombre de secteurs économiques devraient par ailleurs finir sur le long terme par subir le contrecoup de cette décision, avec des difficultés accrues de recrutement d’ici cinq à dix ans. Madame la secrétaire d’État, vous connaissez aussi bien que nous la situation dramatique dans laquelle se trouvent les jeunes pour accéder au marché du travail. L’évolution du financement de l’apprentissage devrait faire l’objet d’une concertation avec les présidents des chambres consulaires, eux qui connaissent les besoins des territoires. Ma question est simple : quelles sont les perspectives du Gouvernement sur l’apprentissage, et comment compte-t-il amortir la demande croissante de ce type de contrats tout en en réduisant les financements ? La parole

l’emploi : sept jeunes sur dix dans les six mois qui suivent la diplomation. Cela ne fait donc aucun doute : l’apprentissage est une solution efficace et concrète pour favoriser l’insertion des jeunes et pour répondre aux tensions de recrutement que rencontrent de nombreuses entreprises. Pour cela, l’État, son opérateur France Compétences, veille à réguler les niveaux de financement de l’apprentissage. Notre objectif est simple : garantir un juste niveau de financement tout en prévenant le risque de marges excessives. Or nous avons constaté l’existence d’écarts encore importants, pour certaines certifications, entre les niveaux de prise en charge et les coûts réels de formation observés dans les CFA. La baisse des niveaux de prise en charge s’inscrit donc dans une démarche de fixation du juste prix, tout en permettant aux CFA de disposer des moyens nécessaires à leur fonctionnement. La ministre déléguée chargée de l’enseignement et de la formation professionnels ouvrira avant la fin de l’année une large consultation avec les partenaires sociaux et les représentants de CFA pour identifier les pistes de simplification et d’amélioration de notre système de régulation

Le permis bateau, contrairement à une idée reçue, n’est pas qu’un objet de loisirs. C’est aussi un préalable nécessaire pour l’accès à de nombreux emplois maritimes : sapeurs-pompiers, pêcheurs, techniciens des ouvrages portuaires, encadrants des activités aquatiques, maîtres-nageurs,

Par ailleurs, les permis voiture, remorque ou moto ont été réintégrés au CPF. Cette absence du permis bateau comme formation éligible dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) pénalise lourdement les potentiels bénéficiaires, qui ne peuvent s’inscrire à ces parcours de formation pourtant particulièrement nécessaires pour accéder à ces métiers de la mer.

maintenant deux mois. En premier lieu, nous devons faciliter l’obtention du permis de conduire. C’est un enjeu d’égalité des chances et d’égalité territoriale. La préparation à l’épreuve du permis de conduire B est ainsi la première certification demandée dans le cadre du CPF depuis 2021, y compris par les demandeurs d’emploi

Les permis permettant de conduire un bateau ne sont toutefois pas éligibles au CPF, car ils ne sont pas considérés comme un prérequis à l’insertion professionnelle dans les zones dans lesquelles les disparités en matière d’accès à la mobilité persistent. Il en est de même pour les brevets ou licences de pilote privé d’avion ou d’hélicoptère. Par ailleurs, si le permis bateau constitue dans un certain nombre de cas, comme vous l’avez rappelé, un prérequis pour l’exercice par le salarié de son emploi, alors il revient à l’employeur, dans le cadre du plan de développement des compétences, de lui proposer des formations d’adaptation à son poste de travail. S’agissant de l’extension à venir, un décret pris en concertation avec les partenaires sociaux doit encadrer cette mesure, car il ne peut pas s’agir d’une extension inconditionnelle. Rappelons que le financement des droits CPF repose sur la contribution directe des employeurs. C’est pourquoi nous devons être vigilants pour que ces droits ne puissent pas être utilisés à d’autres fins que le développement des compétences et la sécurisation du parcours professionnel du titulaire du compte. La

à Mme la ministre de la culture. Dans le cadre de la préparation des jeux Olympiques de Paris 2024, les 250 bouquinistes des quais de Seine ont appris, de la maire de Paris, puis du préfet de police, que l’enlèvement de leurs emblématiques boîtes vertes était indispensable pour la bonne tenue de la cérémonie d’ouverture des jeux Olympiques et des questions de sécurité. Immédiatement, une mobilisation s’est organisée pour que cette décision unilatérale puisse être reconsidérée.

Et le nôtre ! … mais aussi du monde de la culture, et même des Immortels de l’Académie française. En revanche, curieusement, pas de réaction médiatique du ministère de la culture sur la situation des bouquinistes,

Dans le cadre de la sécurisation par l’État de la cérémonie d’ouverture olympique du 26 juillet 2024, la question du retrait temporaire des boîtes des bouquinistes concernés par les périmètres de sécurité se pose.

Lors de cette réunion a été acté le fait que des tests seraient conduits pour déterminer le temps de montage et de démontage des boîtes. Le préfet de police s’est engagé à réétudier finement le linéaire de la cérémonie d’ouverture afin de ne retirer que les boîtes dont le retrait : strictement – nécessaire pour assurer la sécurité des spectateurs. Sa décision dépendra de la capacité réelle à déposer, puis reposer les boîtes dans un délai raisonnable. Les échanges vont se poursuivre à l’aune de ces travaux et de nouvelles réunions seront organisées dans les prochaines semaines. La ministre de la culture restera attentive aux solutions, sûres et positives pour tous, qui pourront être trouvées. Elle reste très attachée aux bouquinistes des quais de Paris, inscrits à l’inventaire national du patrimoine culturel immatériel.

Les chiffres sont édifiants : en un an, 100 000 nouvelles demandes ont été déposées, portant à 2,3 millions le nombre total de ménages en attente d’un logement social. social. Dans le même temps, la production de logements sociaux diminue : il y a eu moins de 100 000 agréments en 2022, alors que 120 000 étaient prévus. Chacun le sait, la baisse des moyens des organismes d’HLM impacte nécessairement la production de ces logements. Tout cela s’inscrit dans une période très tendue où l’augmentation des taux d’intérêt, couplée à la hausse des coûts de la construction, ainsi que la baisse du nombre de logements dans le parc privé entraînent un report de la demande sur le logement social. Néanmoins, la puissance publique a aussi une grande part de responsabilité : ses décisions ont produit des effets négatifs, notamment avec la baisse des aides personnalisées au logement (APL), obligeant les bailleurs à réduire leurs loyers et, de ce fait, à baisser leurs recettes au détriment de leurs capacités d’investissement et de construction.

le logement a été un véritable angle mort des politiques publiques. Madame la secrétaire d’État, pouvez-vous nous détailler les mesures concrètes que le Gouvernement entend prendre afin que les collectivités ne se retrouvent pas en première ligne pour pallier les carences de l’État en matière de logement social ?

face à une crise multifactorielle, le Gouvernement propose une réponse multifactorielle. Contrairement à ce que vous semblez considérer, il n’existe pas de mesure miracle quand une industrie très cyclique est soumise à une multiplication par trois des taux d’intérêt. En revanche, il existe une politique claire : proposer aux Français et aux Françaises des logements de qualité, abordables, qui répondent à leurs besoins et qui soient à proximité des lieux d’emploi. Et pour cela, oui, il faut que les collectivités locales s’impliquent. C’est pour cela que le Gouvernement proposera une réforme de décentralisation qui donnera des moyens et des responsabilités aux collectivités. Dans l’intervalle, le Gouvernement agit. Pour les Français qui travaillent, pour les jeunes, nous voulons développer le logement locatif intermédiaire qui donne accès à des logements à loyers décotés proches des transports dans les villes, grandes ou moyennes. Nous maintenons le prêt à taux zéro, nous facilitons l’accès au crédit, nous développons l’accession sociale. Et pour les Français qui ont besoin d’un logement à un loyer abordable, nous augmentons la capacité d’investissement des bailleurs sociaux. Après la limitation du taux du livret A à 3 %, qui évite une charge de 1,4 milliard d’euros pour les bailleurs sociaux, mon collègue Patrice Vergriete, ministre délégué chargé du logement, a signé avec l’ensemble du mouvement HLM un document d’engagements qui prévoit 1,2 milliard d’euros sur trois ans pour rénover près de 400 000 logements sociaux. Il prévoit aussi 650 millions d’euros de bonifications d’intérêt pour 8 milliards d’euros de prêts. Le Gouvernement est conscient de l’ampleur de la crise de la crise : face à la multiplicité des attentes, il choisit résolument la multiplicité des réponses et la confiance aux collectivités locales, sans dogmatisme et avec pragmatisme. La parole

Ma question se fonde sur l’exemple concret de la communauté de communes de la Vallée de Kaysersberg dans le Haut-Rhin. Cette intercommunalité dispose d’un fonds de concours alimenté par l’indemnité transactionnelle de résiliation de la concession hydroélectrique du lac Noir perçue en 2021. D’un montant de 1,2 million d’euros, alloué jusqu’en 2025, ce fonds vise à financer des projets en lien avec la transition écologique et énergétique, permettant de compenser pour partie la perte de production d’énergie renouvelable sur le territoire. fait face à une difficulté, puisque le code général des collectivités territoriales dispose que « le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assuré, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours ». Alors qu’elle dispose, au travers de ce fonds de concours, de moyens significatifs, la capacité de la communauté de communes de la Vallée de Kaysersberg reste limitée à la capacité financière de ses communes membres, qui sont tenues d’investir à la même hauteur que Conformément aux dispositions législatives en vigueur, les services de l’État ne disposent pas du pouvoir de dérogation dans ce cas spécifique malgré l’intérêt général évident et la pertinence de la démarche vis-à-vis de l’impératif de sobriété que nous partageons largement sur ces travées. Par conséquent, madame la secrétaire d’État, le Gouvernement est-il prêt à envisager une évolution des règles relatives au recours à ce fonds de concours, notamment lorsque celui-ci est mobilisé en faveur de projets visant à favoriser la transition écologique ?

qui détiennent une compétence donnée doivent être en mesure de rester pleinement responsables de la gestion des moyens associés. À ce titre, les fonds de concours constituent déjà un mécanisme visant à assouplir le principe selon lequel la commune et l’intercommunalité concernées restent responsables, chacune, du financement des moyens nécessaires à l’exercice de leurs compétences. La première dérogation à ce principe est l’existence même des fonds de concours entre une commune et son intercommunalité. C’est pourquoi il a été plafonné à un montant qui est celui que la commune finance elle-même. Une dérogation temporaire à ce plafond a été prévue pour les travaux de réparation des biens endommagés lors des violences urbaines de l’été dernier. Aller plus loin, comme vous le suggérez, conduirait à remettre en cause plus largement le principe du financement de la compétence par la commune ou par le groupement qui la détient. Cela n’empêche pas de trouver des solutions pour mobiliser toutes les ressources des territoires en faveur de la transition écologique et énergétique. Il est ainsi possible pour les territoires d’accroître les efforts en matière de coopération, de mutualisation, voire de péréquation, en particulier l’ingénierie technique ou financière nécessaire pour programmer et engager les travaux de rénovation énergétique des bâtiments publics. La parole

Je souhaite attirer l’attention du Gouvernement sur la répartition géographique et financière du fonds vert et du plan d’action pour une gestion résiliente et concertée de l’eau dans les Bouches-du-Rhône. Le changement climatique est là. La prise en compte nécessaire, mais tardive, de ce phénomène s’est notamment traduite par la création du fonds vert, annoncée le 27 août 2022, dont l’objectif est d’accélérer la transition écologique dans les territoires. Dans le cadre de ce plan d’aide, 2 milliards d’euros de crédits déconcentrés aux préfets sont prévus pour soutenir les projets des collectivités et de leurs partenaires publics ou privés, dont 157

je souhaite savoir si le Gouvernement pense mettre à disposition de telles données, car certaines communes volontaires, comme la ville d’Arles, ne semblent pas en être bénéficiaires, alors même que l’urgence des enjeux locaux et la spécificité des sites sont bien présentes. La ville a par exemple prévu un budget annuel de 5 millions d’euros pour la rénovation des canalisations.

de bienvenue. La raréfaction des ressources en eau pose un impératif de sobriété de tous les usages auquel le plan eau, annoncé par le Président de la République le 30 mars dernier, entend répondre, en mobilisant tous les usagers pour atteindre collectivement une baisse de 10 % des prélèvements d’ici à 2030. La lutte contre les fuites dans les réseaux d’eau potable et la réparation des infrastructures et des canalisations sont l’un des leviers pour atteindre cet objectif. L’été 2022 a mis en exergue les fragilités d’alimentation en eau potable d’un nombre important de communes. Le plan eau en tire les avec 180 millions d’euros par an prévus pour réduire les fuites et sécuriser l’approvisionnement en eau potable. Ces moyens doivent permettre d’intervenir de manière ciblée en soutien des collectivités structurellement fragiles, là où un juste prix de l’eau et la solidarité intercommunale ne suffisent pas à assurer le renouvellement patrimonial. L’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse a financé depuis 2019 des actions d’amélioration de la qualité du service d’eau potable à hauteur de 290,4 millions d’euros, ainsi que des actions de protection de la ressource à hauteur de 25,6 millions d’euros. Elle bénéficiera dès 2024 d’une quote-part des 180 millions, que je viens d’évoquer, pour renforcer son action selon les priorités et conditions d’éligibilité définies dans son programme d’intervention arrêté par son conseil d’administration après avis conforme du comité de bassin. La parole

L’urgence, que nous partageons, est la définition de mesures concrètes permettant de mieux protéger les riverains des nuisances, tout en tenant compte d’hypothèses réalistes de développement de l’aéroport. Avec l’approbation, en juin, du plan de prévention du bruit dans l’environnement de l’aéroport, les conditions étaient réunies pour lancer une étude d’impact.

S’agissant de l’objectif de généralisation des descentes continues, je vous confirme que c’est l’une des priorités du ministre pour réduire les émissions de CO2 et les nuisances sonores. de ce type entraînerait des effets de redistribution importants. Ainsi, comme Clément Beaune a pu le préciser aux élus et représentants des riverains reçus le 9 mai dernier, il a été décidé de tirer parti des consultations en cours s’agissant de l’aéroport d’Orly. Les évolutions possibles concernant Charles-de-Gaulle pourront être rediscutées ; en parallèle, les services de l’aviation civile travaillent à l’amélioration du taux de descentes continues. Je vous confirme, enfin, que le Gouvernement est très attaché aux politiques publiques de lutte contre les nuisances sonores aériennes, tout particulièrement en région parisienne, où la densité de population rend la question particulièrement

ainsi que de l’article L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales. Ils préfèrent généralement solliciter les forces de l’ordre ou le procureur de la République, mais il existe certaines situations dans lesquelles leur intervention est à la fois indispensable et préférable.

par l’article L. 330-2 du code de la route. Et le législateur a bien fait : cette faculté permet aux maires, en tant qu’OPJ, de veiller sur l’ordre public, en identifiant les auteurs de certaines infractions, routières ou pénales, tout en conservant la faculté d’adapter la réponse à y apporter, depuis une simple discussion jusqu’à un rappel à la loi, voire une transmission au procureur de la République.

Ce pouvoir est d’autant plus important qu’il contribue à consolider l’autorité des maires dans leur commune, dont nous savons qu’elle est parfois durement éprouvée. Malgré ces raisons, le pouvoir réglementaire n’est pas encore intervenu afin d’expliciter et de préciser les conditions d’accès des maires au système d’immatriculation des véhicules. Madame la secrétaire d’État, les maires peuvent-ils compter sur votre intervention pour y remédier ? La

immatriculés en France. Il répond à des enjeux importants, notamment pour la sécurité routière et la lutte contre la criminalité. Ce système, qui comporte des données à caractère personnel, est soumis aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi qu’au règlement général sur la protection des données L’accès aux données est donc autorisé en fonction de la finalité recherchée, sous le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), et fait l’objet d’une traçabilité. Ainsi, en application de l’article R. 330-2 du code de la route, le maire bénéficie d’un accès direct aux informations du SIV dès lors que cet accès s’inscrit dans le cadre des attributions prévues par le code de l’environnement aux seules fins d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation. Cela concerne le cas, par exemple, d’un véhicule épave stocké sur la voie publique, privé des éléments indispensables à son utilisation normale et non susceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols. L’article L. 330-2 du code de la route donne également accès au SIV aux maires et à leurs adjoints en tant qu’officiers de police judiciaire dans l’exercice des missions de police judiciaire et sous l’autorité du procureur de la République. Afin de pouvoir bénéficier de cet accès, qui ne peut être délégué, les maires doivent se rapprocher des services préfectoraux, habilités à gérer les accès au système d’immatriculation des véhicules. Ces accès restent soumis à des exigences techniques visant à assurer la sécurité

En effet, l’arrêté du 22 juillet 2023 portant sur cette reconnaissance a engendré dans mon département incompréhension et colère parmi les élus et citoyens des communes concernées. déposés dans le Tarn-et-Garonne, seulement six communes ont obtenu cette reconnaissance, apparemment en raison du non-respect du critère météorologique mentionné dans une circulaire au nom barbare. Vous conviendrez que cette réponse n’est pas acceptable. Cette situation est d’autant plus déconcertante que certaines communes de Lot-et-Garonne, distantes de quelques centaines de mètres seulement, ont été classées, quant à elles, en état de catastrophe naturelle. La frustration et la colère montent parmi les élus locaux et la population. Une colère que je partage, car une simple visite sur le terrain suffit pour constater les impacts de la sécheresse sur les habitations. J’ai eu moi-même l’occasion de le constater lors de mes déplacements. Comment expliquer qu’un habitant de Léojac ou de La Salvetat-Belmontet puisse déposer à sa compagnie d’assurances un dossier d’indemnisation, alors que celui de Génébrières, commune située à quelques mètres de là, ne le puisse pas, comme si la sécheresse s’était arrêtée au panneau d’entrée du village ? Je pourrais vous donner de multiples exemples de cette nature. Madame la secrétaire d’État, pourriez-vous nous fournir des clarifications sur les critères ayant mené à ces décisions et nous expliquer les raisons de ces évidentes disparités entre des communes géographiquement si proches ? Une modification de l’arrêté du 22 juillet est-elle envisageable ? De plus, dans un esprit de transparence et de confiance avec les citoyens et les élus locaux, quelles actions concrètes le Gouvernement envisage-t-il de mettre en place pour rendre le processus de classement en état de catastrophe naturelle plus clair et compréhensible par tous ?

L’épisode de sécheresse et de réhydratation des sols de 2022 a été particulièrement sévère et a donné lieu au dépôt d’un nombre record de demandes communales de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle – il y en Sur ces demandes, 6 313 ont reçu une suite favorable pour un montant d’indemnisation évalué à plus de 3 milliards d’euros. Dans le Tarn-et-Garonne, sur les 152 demandes communales déposées, 69 ont fait l’objet d’une suite favorable. La reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle n’intervient que lorsque les épisodes de sécheresse présentent une intensité anormale avérée au regard des critères de la circulaire du 10 mai 2019. Les données mobilisées pour instruire les demandes sont suffisamment précises pour permettre une analyse de l’intensité des épisodes de sécheresse propre à chaque territoire communal. Par ailleurs, au-delà de la motivation des décisions, qui est désormais directement précisée dans les arrêtés interministériels, des documents explicatifs propres à la situation de chaque commune sont transmis

a réuni plus de 40 000 personnes et quelque 20 000 véhicules et caravanes, sur une commune de 603 habitants. Il s’est déroulé du 3 au 10 septembre 2023 sur autorisation de Mme la Première ministre, sans concertation et au mépris des élus locaux. Pourtant, en 2017, le Premier ministre, M. Édouard Philippe, avait engagé la parole de l’État sur la position inverse, tant les nuisances et perturbations avaient été insupportables pour les habitants, et les dommages générés par ce rassemblement considérables et fort peu indemnisés. Les élus locaux sont inquiets pour l’année prochaine. Le maire de la commune mosellane de Suisse a même démissionné face à la colère de la population et des agriculteurs. le caractère manifestement inadapté de la base de Grostenquin pour l’accueil du rassemblement « Vie et Lumière » ne laisse planer aucun doute. Cette année encore, force est de constater que le droit à la tranquillité à la salubrité publiques a été nié aux habitants des communes rurales concernées. Outre les problèmes d’hygiène, d’aménagement du territoire et d’organisation de la voie publique, que penser du rationnement de l’eau potable imposé aux quelque 1 800 habitants des communes de Bistroff, Guessling-Hémering et Grostenquin pendant plus de sept jours, alors que, dans le même temps, les gens du voyage se permettaient d’utiliser cette eau, mise à leur disposition par les collectivités, pour – excusez du peu ! – laver leurs véhicules et remplir leurs piscines privatives ? Ces troubles excessifs et ces abus, nous les connaissions et vous les connaissiez, puisque le Premier ministre

Je tiens également à souligner le caractère constructif du dialogue mené avec l’association Vie et Lumière. Je tiens ensuite et surtout à rectifier certaines de vos affirmations. Premièrement, ce rassemblement n’a pas compté 40 000 participants ; ils étaient entre 20 000 et 25 000. Plus ! Deuxièmement, les habitants des communes de Bistroff, Guessling-Hémering et Grostenquin n’ont pas subi de restrictions d’accès à l’eau. Le débit d’eau fourni à l’organisateur de

ont donc uniquement concerné les gens du voyage : le préfet de la Moselle n’a pas rationné l’alimentation en eau des habitants des communes limitrophes ! Troisièmement, il convient de rappeler que le régime applicable en matière de stationnement des gens du voyage est déterminé par la loi du 5 juillet 2000 Cette loi ne fait pas primer les droits des gens du voyage sur les principes fondamentaux de la République, mais établit un équilibre entre leur aspiration à pouvoir stationner dans des conditions décentes, d’une part, et le souci d’éviter des installations illicites, En cas de méconnaissance des règles établies, le préfet peut faire usage de ses pouvoirs de police. Des poursuites judiciaires peuvent également être engagées. À cet égard, l’organisation de déplacements de la gendarmerie sur le site, au contact des élus locaux, a permis de faciliter et d’accélérer l’enregistrement des plaintes déposées pour chaque dégradation constatée. Enfin, pour l’avenir, le cabinet du ministre de l’intérieur et des outre-mer rencontrera prochainement les représentants de cette association, afin de préparer les prochains événements et de réfléchir à une diversification des lieux d’accueil des grands rassemblements. La parole est à M. Claude Nougein,

payée par l’employeur le plus important des quatre dernières années. C’est donc la collectivité qui doit verser ladite indemnité, alors même que la personne a démissionné ! C’est une véritable prise en otage des collectivités territoriales, qui sont de plus en plus contraintes dans leur budget, en particulier les petites communes rurales. Plusieurs exemples se sont multipliés cette année dans mon département de Corrèze. Par exemple, un agent a occupé un poste en CDD, qui est devenu vacant ; cet agent aurait donc pu renouveler son CDD. De plus, l’agent en question demande également à intégrer dans son ARE une prime d’assiduité obtenue pendant ces six mois d’activité dans le privé, prime témoignant de sa capacité à occuper cet emploi. emploi. Cet agent avait plus de vingt ans d’ancienneté dans le poste communal ; compte tenu de son âge, la durée d’indemnisation pourrait excéder trois ans, en attendant la liquidation de ses droits à la retraite.

Dans le cas de figure décrit ici, l’agent titulaire bénéficie donc à la fois de la garantie de l’emploi et de l’indemnisation du chômage. Par rapport au secteur privé, c’est complètement ubuesque ! Les deux dispositifs se cumulent, ce qui n’est pas dans l’esprit du statut de fonctionnaire

le versement de l’allocation de chômage est notamment conditionné au caractère involontaire de la perte d’emploi. À cet égard, le règlement d’assurance chômage précise que la fin d’un contrat à durée déterminée constitue une privation involontaire d’emploi. En outre, le code du travail prévoit que l’employeur territorial est débiteur de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Ce sont les agents de Pôle emploi qui doivent ensuite procéder au contrôle de la recherche effective d’emploi qui conditionne le versement de l’ARE. Enfin, la lecture combinée des articles L. 2321-2 et R. 2321-2 du code général des collectivités territoriales autorise le provisionnement pour risques et charges dès l’apparition d’un risque avéré. Les employeurs territoriaux en auto-assurance étant tenus de supporter la charge de l’indemnisation du chômage de leurs anciens fonctionnaires, il leur appartient d’estimer le risque et, le cas échéant, de le provisionner. Le Gouvernement considère que tout autre dispositif visant à financer cette dépense sur d’autres fonds, notamment par une mutualisation du risque, induirait nécessairement une charge financière supplémentaire pour les employeurs, alors même que ces situations restent peu nombreuses. La parole

le myélome multiple, cancer de la moelle osseuse, est une maladie rare qui touche chaque année près de 5 400 nouvelles personnes. Cette grave pathologie affecte, au total, 30 000 personnes en France. Si les traitements ont évolué et permettent à certains patients de vivre avec la maladie, des formes plus agressives rendent inefficaces les traitements proposés en France. L’Agence européenne des médicaments a délivré des autorisations de mise sur le marché européen

Or la Haute Autorité de santé (HAS), chargée en France de l’évaluation de ces médicaments innovants, n’accorde pas d’autorisation de mise sur le marché. Ce refus s’appuie sur une doctrine comparative Pour l’Association française des malades du myélome multiple, cette décision n’est pas acceptable, car d’autres pays européens disposent de ces médicaments qui ont montré des résultats encourageants. Faute d’accès à ces traitements, les malades en échec thérapeutique, déclarés réfractaires après administration des traitements actuellement autorisés en France, sont condamnés à une mort certaine.

Ces spécialités ont bénéficié d’autorisations de mise sur le marché conditionnelles délivrées par la Commission européenne à un stade précoce de leur développement. Sur la base de la reconnaissance d’une présomption d’innovation et en l’absence de traitements appropriés, la HAS a délivré une autorisation d’accès précoce à ces trois spécialités. Cette procédure dérogatoire exceptionnelle a permis à des patients français, en impasse thérapeutique, de bénéficier de ces traitements de façon anticipée.

de leur développement, la HAS a fait évoluer sa doctrine en février 2023. La nouvelle approche proposée repose sur un équilibre entre développement clinique accéléré et maîtrise du niveau d’incertitudes, au bénéfice des patients.

multiple en rechute et réfractaire ayant reçu au moins trois traitements antérieurs. Concernant la spécialité Carvykti, le laboratoire a fait le choix de retirer sa demande de prise en charge dans le cadre d’un remboursement par l’assurance maladie. Enfin, s’agissant de la spécialité Tecvayli, l’autorisation d’accès précoce est toujours en cours. Par ailleurs, dans le cadre du plan France 2030, le volet « Biothérapies et Bioproduction de thérapies innovantes » des programmes et équipements prioritaires de recherche (PEPR) répond enfin à l’enjeu de développement de ce type de thérapie. La parole

que la France, qui a des hématologues et des spécialistes du myélome extrêmement brillants et professionnels, puisse avancer beaucoup plus rapidement, au moins à la vitesse de l’Europe : ce serait une

de laquelle les collectivités devaient se mettre en conformité. En résumé, là où le législateur avait instauré une possibilité pour les élus, le décret d’application a transformé cette faculté en obligation, donc en contrainte. Madame la secrétaire

Le décret du 6 décembre 2022 est venu préciser les modalités d’application de cet article. Lors de l’examen de ce texte, le Conseil d’État a été particulièrement attentif aux garanties d’indépendance et d’impartialité des personnes physiques pouvant être désignées pour assurer ces fonctions. Le décret dispose que l’organe délibérant de chaque collectivité territoriale, groupement de collectivités territoriales ou syndicat mixte désigne le référent déontologue : soit une ou plusieurs personnes, soit un collège. Le texte permet également la désignation d’un même référent déontologue de l’élu local par plusieurs collectivités, groupements de collectivités ou syndicats mixtes, par délibérations concordantes. Il n’existe pas de possibilité de mutualisation, mais il est possible de désigner le même référent ou collège ; par exemple, un conseil départemental, une communauté de communes et des communes non-membres de cette communauté

et, de manière générale, sur les inégalités d’accès à l’offre de soins. Encore récemment, le départ imprévu d’un médecin est venu fragiliser l’unité de soins intensifs et spécialisés pour enfants et adolescents (Usisea) du centre hospitalier de Laval, alors même que son équipe de pédopsychiatrie doit gérer l’ensemble des consultations sur le territoire mayennais, dans cette unité comme dans les centres médico-psychologiques et dans le service de suivi à domicile. Notons que cette unité de soins intensifs permet l’hospitalisation complète des enfants ayant des troubles psychiatriques lourds. Or, aujourd’hui, ce service ne compte plus que quatre contre dix auparavant. De jeunes patients en grande souffrance occupent donc des lits qui ne leur sont pas destinés ; d’autres attendent leur hospitalisation, parfois pendant plus de dix-huit mois. Dans ce contexte, les familles sont extrêmement inquiètes pour leurs enfants

L’ARS a annoncé hier un plan global d’urgence : une enveloppe de 1 million d’euros, dont plus de 600 000 euros pour la pédopsychiatrie, aurait été débloquée. Ces crédits doivent permettre de recruter une dizaine de soignants afin de renforcer les équipes. C’est une bonne nouvelle, mais il reste encore beaucoup à faire. Aussi, madame la secrétaire d’État, alors que la santé mentale et psychique des jeunes représente un enjeu particulièrement important après la crise sanitaire, je souhaite connaître les intentions du Gouvernement pour maintenir un accès aux soins pédopsychiatriques durable et équitable en Mayenne. La parole

Conscients de l’urgence de la situation, nous nous sommes engagés dès le début du mois aux côtés des équipes médicales pour proposer un plan global d’urgence. Son objectif Son objectif est de sécuriser la prise en charge des patients, d’augmenter la capacité à répondre aux demandes de consultations dans les centres médico-psychologiques et de redonner des perspectives aux acteurs de terrain.

la création d’un hôpital de jour pour les adolescents de 15 ans à 18 ans sur le site du centre hospitalier de Laval, avec une capacité de cinq places dès 2023 et une cible de dix places en 2025 troisièmement, le renforcement de l’offre ambulatoire de pédopsychiatrie dans le département, dans les centres médico-psychologiques actuels, mais aussi par un élargissement du dispositif Escapad sur le département. En lien avec l’ARS des Pays de la Loire, nous avons mobilisé une enveloppe de 1 million d’euros, dont 600 000 euros pour la pédopsychiatrie, enveloppe qui sera consacrée à l’accompagnement de l’ensemble de ces mesures. Ces crédits permettront notamment le recrutement sans délai de plus de dix soignants pour venir renforcer l’ensemble des équipes sur le territoire. La parole

du système de santé sur notre territoire. On ne compte plus les fermetures de services dans nos établissements, de celle du service de médecine à l’hôpital de La Charité-sur-Loire à celle du centre périnatal de proximité de Cosne-sur-Loire, en plus de celle de la maternité d’Autun.

sans nier les difficultés réelles que vous évoquez, le Gouvernement est pleinement mobilisé pour renforcer l’accès aux soins dans la Nièvre. Ce département n’est pas laissé à l’abandon, comme vous le suggérez Au contraire, nous mobilisons tous les leviers pour accroître l’attractivité de ce territoire, en lien avec l’ensemble des parties prenantes. Pour maintenir une offre de soins sur le secteur de Château-Chinon, nous avons travaillé, en lien avec les pouvoirs publics locaux, à la mise en place de consultations de soins non programmés ; elles sont effectives depuis le 4 septembre. Dans le cadre du Ségur de la santé, nous soutenons également la reconstruction de l’hôpital de Cosne-sur-Loire, qui permettra d’offrir aux professionnels de santé un outil de travail moderne attractif pour de nouveaux médecins. Dans les centres hospitaliers du département, la réserve sanitaire a été activement mobilisée pour accompagner les établissements, avec une soixantaine de missions réalisées, et éviter les fermetures de lits. En outre, nous travaillons activement à l’élaboration d’un plan pluriannuel territorial qui s’emploiera à soutenir toute forme de dispositifs allant de la formation à l’emploi et à la fidélisation des professionnels de santé. Par ailleurs, nous mobilisons une enveloppe de 2 millions d’euros supplémentaires pour financer les projets en faveur de l’attractivité dans la région Bourgogne-Franche-Comté Bourgogne-Franche-Comté et plus particulièrement dans la Nièvre. Enfin, il faut citer le pacte territoire-santé de la Nièvre, en cours de finalisation, qui concrétise un engagement pour le développement d’une vingtaine d’actions partagées avec le conseil départemental afin de répondre aux thématiques de l’accès aux soins, du bien vieillir et de la santé mentale des jeunes. Vous le voyez, le Gouvernement est pleinement mobilisé. La parole Aujourd’hui, les Nivernais, dont l’espérance de vie est inférieure de deux ans à la moyenne nationale, sont lassés des discours, des concertations et des schémas : ils vous demandent d’agir réellement ! Nous aussi

Lors de la crise sanitaire, des entrepreneurs se sont mobilisés pour réindustrialiser notre pays ; ils ont mis sur pied des lignes de production française de masques sanitaires. À la fin de 2020, la France était autosuffisante, avec une capacité de production de cent millions de masques par semaine. Le problème est que cet effort collectif est aujourd’hui battu en brèche par la commande publique elle-même. Nombre d’établissements publics ont en effet changé de braquet ; ils reproduisent les erreurs du passé en important ces produits stratégiques, laissant nos industriels sans débouchés. À Nersac, dans mon département de la Charente, la ligne de production de l’usine Next Safe est à l’arrêt. Malgré la circulaire de mars 2023 réformant les critères de sélection des appels d’offres, les ministères et les établissements publics s’approvisionnent à l’étranger, se focalisant sur le critère unique du prix au détriment de la qualité technique et logistique, ou encore de la prise en compte

pourtant que le projet de loi relatif à l’industrie verte en accélère la mise en œuvre obligatoire, en la fixant en 2024 au lieu de 2026 pour des produits clés de la décarbonation. Sur le sujet spécifique des produits de santé, des actions fortes sont d’ores et déjà menées pour renforcer les débouchés, en officine et sur les marchés publics hospitaliers, des entreprises qui fabriquent en Europe des médicaments et dispositifs médicaux stratégiques. Ainsi, l’instruction n° 149 de la direction générale de l’offre de soins (DGOS) du 24 mai 2022 incite les acheteurs hospitaliers à intégrer les enjeux de sécurité d’approvisionnement à leur politique d’achat de produits de santé stratégiques, étant entendu qu’une production localisée en Europe est la meilleure garantie de la sécurité d’approvisionnement de nos hôpitaux. L’instruction du 24 mars 2023 de la DGOS va dans le même sens, en demandant explicitement une adaptation du processus d’achat des fournitures, produits de santé et équipements critiques, dont font partie les masques. L’objectif est de valoriser les éléments différenciant positivement les industriels français et européens, dans le respect du droit de la commande publique. Cette instruction retient le principe de la compensation financière, pour les établissements de santé concernés, des surcoûts entre les sources d’approvisionnement européennes sécurisantes et les autres sources. De plus, lorsque la sécurisation des approvisionnements est un enjeu majeur, et sous certaines conditions, l’implantation européenne des moyens de production peut être demandée en application de l’article L. 2112-4 du code de la commande publique.

publics se tournent réellement vers les productions françaises, que les instructions soient enfin appliquées et les sanctions prises en cas de manquement ; sinon, il n’y aura bientôt plus de filière de masque en France, et ce seront alors des centaines de millions d’euros, y compris d’argent public, qui auront été dépensés, et des milliers d’emplois créés, pour rien

est particulièrement dégradée. Un chiffre témoigne de l’urgence à étoffer les effectifs : au tribunal judiciaire, le nombre de dossiers d’information par cabinet de droit commun est de 124, quand le seuil d’alerte est fixé à 72. Le seuil est également amplement dépassé dans les cabinets chargés de la grande criminalité. Bien que le département d’Ille-et-Vilaine connaisse une croissance démographique soutenue et continue depuis 2008, le nombre moyen de juges d’instruction dans le ressort de la cour d’appel de Rennes n’est que de 5,1 pour 1 million d’habitants, quand le ratio national s’élève à 8,4. C’est le plus bas de France… France… Traduit concrètement, cet écart signifie qu’il manque quinze juges d’instruction. Malgré l’investissement des magistrats, les conséquences de cette insuffisance sont réelles. Le stock de dossiers augmente, les délais d’achèvement des procédures sont allongés, le risque de prescription s’accroît. Aujourd’hui, l’ensemble de la chaîne pénale est « embolisée », à l’instar des services d’enquête et des experts auxquels la justice a besoin de recourir. En d’autres termes, la situation de la justice pénale à Rennes a atteint un point critique.

À la cour d’appel, les effectifs ne connaissent aucune vacance. Au sein du tribunal judiciaire de Rennes, les effectifs du service de l’instruction sont également au complet : les trois postes de juge ainsi que les trois postes de vice-président sont pourvus. Par ailleurs, les effectifs globaux du tribunal judiciaire de Rennes connaissent un surnombre de juge non spécialisé. Seul un poste de juge des enfants est vacant, mais il est numériquement compensé par un second surnombre de juge non spécialisé.

bénéficiera à ce titre d’une augmentation sensible de ses effectifs à l’horizon de 2027. Ce sont en effet au moins 58 magistrats, 61 greffiers et 54 attachés de justice supplémentaires qui viendront renforcer les juridictions du ressort de cette cour. Entre 2017 et 2027, ce seront donc plus de 101 magistrats supplémentaires qui seront venus renforcer le ressort de la cour d’appel de Rennes ! Je veux être clair : tous ces renforts prévus dans la loi d’orientation et de des remplacements des départs à la retraite. Dans le cadre de la politique fixée par la Chancellerie – celle de la confiance dans les acteurs de terrain –, il appartient désormais aux chefs de la cour d’appel de Rennes de proposer la répartition de ces effectifs au sein des différentes juridictions de leur ressort en fonction d’une analyse locale, au plus près des besoins. Je vous confirme que ces renforts permettront, le cas échéant, de renforcer les effectifs de juges d’instruction du ressort du tribunal judiciaire de Rennes.

Outre l’identité culturelle qu’il véhicule, cet élevage participe de manière prépondérante à la préservation d’un écosystème et d’une biodiversité uniques au monde : la Camargue.

Ce phénomène touche également les festivités taurines du sud de la France, qui sont organisées par des communes ou des associations. Au cours des dernières années, au regard des difficultés conjoncturelles, nos manadiers ont mené de véritables actions de diversification de leur activité : obtention d’une appellation d’origine protégée (AOP), réception de visiteurs, location de salles, etc. Malgré cela, nos manades risquent aujourd’hui de disparaître définitivement et, avec elles, une part de notre culture, de notre économie locale, mais aussi des acteurs essentiels au maintien d’un écosystème. En effet, la Camargue est un environnement fortement fragilisé. Ma question est donc simple. Monsieur le ministre, que comptez-vous mettre en œuvre pour protéger les manadiers ?

Chaque année, les services de l’État, en lien avec les communes, contribuent à l’organisation des fêtes camarguaises, notamment pour ce qui relève de la sécurité publique. Le Gouvernement est mobilisé pour que chacun – particulier, entreprise, collectivité – puisse bénéficier d’une assurance adaptée aux risques aux risques auxquels il fait face, en contrepartie d’une responsabilisation par une plus grande prévention. À titre d’exemple, le Gouvernement a lancé une mission dédiée à l’assurabilité face au réchauffement climatique, qui rendra ses conclusions en décembre prochain. De la même manière, il lancera prochainement une mission consacrée à l’assurabilité des collectivités territoriales, après les difficultés qu’ont connues les communes touchées par les émeutes de la fin du mois Le Gouvernement veillera ainsi à l’accès à une assurance, dans des conditions de couverture raisonnables, des communes et manadiers organisateurs de fêtes camarguaises. En plus d’une mobilisation des assureurs, le Gouvernement appelle aux efforts de prévention les plus ambitieux possible des organisateurs de ces fêtes, afin de réduire les risques associés et, ainsi, de faciliter leur accès à l’assurance. Les services déconcentrés de l’État pourront aussi être mobilisés dans les efforts tant de prévention que d’accès à l’assurance.

et numérique. Monsieur le ministre, un décret du 25 août dernier élargit à 2 200 nouvelles communes la possibilité de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires était très attendu par de nombreuses communes jusqu’à présent exclues de ce dispositif. Malgré cet élargissement, beaucoup d’entre elles restent oubliées. C’est le cas de Dieppe, de Dieppe, d’Eu, du Tréport ou de Saint-Jouin-Bruneval, près d’Étretat, par exemple, en Seine-Maritime. Rien ne justifie pourtant leur exclusion du dispositif. À Dieppe, les résidences secondaires ont augmenté de 407 % en cinquante

Au Tréport, 490 demandes de logement social sont en souffrance. Eu compte 520 demandes actives. Pour ces communes, augmenter la taxe d’habitation sur les résidences secondaires permettrait d’accéder à de nouvelles recettes, bienvenues dans le contexte d’inflation que nous connaissons. Cette mesure contribuerait aussi à une meilleure maîtrise de l’habitat, face à l’accroissement du nombre des résidences secondaires et des locations de courte durée. Enfin, l’exclusion de certaines communes du dispositif risque de renforcer les problèmes, puisque les acquéreurs de résidences secondaires se porteront plutôt sur les communes exclues du décret que sur les autres, accroissant encore la tension.

cette mesure ? La parole est à M. le ministre délégué. Madame la sénatrice, vous avez appelé mon attention sur les critères qui ont été retenus pour établir, par décret du 25 août 2023, la liste des communes intégrant les zones tendues. Comme vous le savez, ces critères permettent de définir les communes faisant face à des difficultés sérieuses d’accès au logement et pour lesquelles deux dispositifs fiscaux incitatifs frappant la rétention foncière sont applicables : la taxe annuelle sur les logements vacants (TLV) et, sur délibération communale, la majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. La réforme des zones tendues s’est articulée autour de deux axes. Le premier est l’actualisation du périmètre des zones tendues historiques d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants,

dans le parc locatif social. Le second vise à répondre à la forte demande politique dont votre question atteste. Il s’agit de l’élargissement de ces zones aux communes qui, sans appartenir à des zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, présentent une forte tension immobilière résultant notamment d’une proportion élevée élevée de résidences secondaires en plus de niveaux élevés des loyers et des prix d’acquisition des logements anciens. C’est sur le fondement de ces critères et après consultation des associations d’élus locaux, comme le Gouvernement s’y était engagé, qu’une liste actualisée de communes a été établie. La nouvelle liste permet ainsi d’améliorer la prise en compte de la situation particulière des communes touristiques les plus exposées aux difficultés d’accès au logement, en leur confiant les leviers fiscaux pour y répondre. Il s’agit d’un élargissement très sensible, puisque le nombre de communes a été multiplié par trois,

qui est confrontée à un déficit de réseaux internet et mobile en raison de la présence d’une station de radioastronomie. Cette dernière, par crainte d’interférences avec ses travaux scientifiques, refuse l’installation d’un réseau 4G. Cependant, des exemples aux Pays-Bas démontrent que, grâce

que pour le développement économique et scientifique des territoires. La commune de Nançay se trouve ainsi confrontée à un défi majeur, entravant son attractivité et son potentiel de croissance. Je vous invite à étudier de nouveau cette situation et à explorer les possibilités techniques et réglementaires permettant de concilier les exigences de la station de radioastronomie avec les besoins en réseau haut débit de la commune de Nançay. Favoriser le progrès scientifique tout en assurant un accès équitable aux technologies de communication est essentiel. Comment le Gouvernement compte-t-il relever ce défi afin de garantir un développement équilibré et harmonieux de Nançay ? de Nançay ? La parole est à M. le ministre délégué. Monsieur le sénateur, le cas de la commune de Nançay est un cas particulier bien connu des services de l’État. Comme vous l’avez rappelé, cette dernière abrite un observatoire radioastronomique de classe mondiale, notamment le quatrième plus grand radiotélescope à l’échelon mondial. Le principe de fonctionnement des instruments présents sur le site de Nançay repose sur la réception et l’analyse de signaux radioélectriques de faible intensité, émis depuis l’espace par les corps célestes. Ces signaux faibles et naturels sont donc susceptibles d’être perturbés par toute autre émission radioélectrique proche, par exemple celles qui proviennent d’une antenne fournissant un service de communication mobile. Pour limiter ce type de risque, une zone de servitude radioélectrique a été établie par un décret du 8 décembre 2010. interdit le déploiement d’équipements radioélectriques de nature à perturber le bon fonctionnement des équipements déployés par l’observatoire dans une zone proche de celui-ci, incluant la commune de Nançay. Il en résulte en effet une difficulté

avec celui de Nançay, n’apparaît pas directement transposable à la situation qui nous préoccupe : le site en question déploie des technologies différentes en termes tant d’équipements que de fréquences. Je souhaite néanmoins que toutes les solutions techniques puissent être envisagées. C’est à ce titre que le Gouvernement a demandé aux services de Bercy et à l’Agence nationale des fréquences de travailler, en lien avec les préfectures concernées, l’Autorité de régulation des à l’examen des options conciliant les contraintes de chacune des deux parties et à l’identification, le cas échéant, des conditions et des scénarios de leur mise en œuvre. J’espère que ces travaux pourront aboutir à une expérimentation et à des propositions concrètes dans le courant de l’année 2024,

Monsieur le ministre, de plus en plus de communes et d’intercommunalités, petites ou grandes, rurales comme urbaines, rencontrent des difficultés dans leur recherche d’un prestataire d’assurance pour couvrir les risques auxquels elles sont confrontées. Bien souvent, les prestataires ne répondent pas aux appels d’offres et, quand ils le font, un grand nombre d’entre eux proposent des tarifs très élevés, difficilement supportables pour des budgets communaux ou intercommunaux. De nombreux maires et présidents d’intercommunalité se retrouvent donc dans l’incapacité de souscrire un contrat d’assurance, ce qui les laisse seuls face aux risques et, surtout, face aux conséquences susceptibles d’entraver le bon fonctionnement des services publics locaux. de mars dernier, Mme la ministre chargée des collectivités territoriales a répondu à mon collègue Didier Marie que le Gouvernement avait pleinement conscience de ces difficultés ; elle s’était engagée à revenir vers lui. Récemment, M. le ministre de l’économie et des finances a annoncé des mesures pour faire face au problème, notamment la possibilité pour les collectivités de saisir le médiateur de l’assurance. Je ne suis pas certaine que cela rassure les maires et présidents d’intercommunalité concernés. En revanche, la proposition de lancer une mission associant experts, élus et assureurs, afin de définir des solutions de long terme

par les récentes violences urbaines de l’été 2023, dont le coût assurantiel s’élève à près de 200 millions d’euros pour les dommages aux biens des collectivités territoriales. Je rappelle qu’environ 500 collectivités ont été touchées. Dans l’immédiat et afin de contribuer à l’instauration d’un climat de confiance entre les collectivités territoriales et les assureurs, le Gouvernement a annoncé à la fin du mois de septembre dernier la conclusion d’un accord avec les assureurs, afin que ces derniers mettent en place le recours à la médiation de l’assurance, intervenant comme un médiateur conventionnel, pour les litiges portant sur les contrats d’assurance des collectivités territoriales.

des conventions fiscales internationales avec des pays à haute capacité contributive – notamment l’Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats arabes unis. En l’espèce, c’est un peu comme dans le sketch de Coluche : plus on peut payer, moins on paye

permettent de prévenir les doubles impositions auxquelles seraient sinon confrontés nos entreprises et nos concitoyens, en particulier ceux qui résident à l’étranger, pour un même revenu perçu. Elles remplissent également un objectif économique important, offrant un cadre juridique sécurisé aussi bien pour ceux qui investissent en France que pour nos entreprises qui investissent hors de France. Les conventions servent aussi à mettre en œuvre des dispositifs essentiels pour que nos administrations puissent lutter contre la fraude. Je pense en particulier aux clauses qui nous permettent d’échanger des renseignements fiscaux et, dans certains cas, d’obtenir que nos partenaires nous assistent pour le recouvrement de nos créances. Établir les gains et les coûts budgétaires d’une convention en particulier est impossible

si cette absence devait dissuader les investissements, donc les flux imposés. Chaque convention contient de nombreuses clauses différentes et est le fruit d’une négociation avec un autre État, qui a lui-même des intérêts à faire valoir. Les conventions que vous mentionnez, celles qui nous lient aux États du Golfe et qui sont négociées, conclues et ratifiées par le Parlement en leur temps, n’ont pas échappé à cette règle. Nos services s’emploient bien entendu à moderniser progressivement ce réseau conventionnel, mais c’est une entreprise longue et qui suppose la même volonté chez nos partenaires. Ils s’emploient aussi à faire avancer certains chantiers pour plus robustes certaines règles de fiscalité internationale, notamment en matière de risques d’optimisation. Ainsi, la mise en œuvre du chantier (Beps) de l’OCDE contribue à apporter une réponse, au travers de la modernisation de nos conventions bilatérales par l’instrument multilatéral que nous avons ratifié en 2018. 2018. Il prévoit plusieurs clauses anti-abus, notamment pour éviter le. Cet instrument, s’il est ratifié par les deux États parties à une convention bilatérale, modifie cette dernière. C’est le cas par exemple pour l’Arabie saoudite, Bahreïn, les Émirats arabes unis ou encore Oman.

des affaires étrangères. Monsieur le ministre, je vous interpelle aujourd’hui au sujet du droit à la retraite de nos compatriotes établis en Nouvelle-Zélande. Le système de retraite néo-zélandais prévoit l’octroi d’un montant de base universel auquel sont éligibles les citoyens néo-zélandais, ainsi que les étrangers établis dans ce pays. Cette pension financée par l’État interdit le cumul de la retraite d’État néo-zélandaise avec une pension de retraite provenant de l’étranger. Ainsi, nos compatriotes ayant eu une carrière dans les deux pays reçoivent une retraite néo-zélandaise défalquée du montant qu’ils perçoivent de France. en résulte des situations de précarité et une profonde injustice pour nos compatriotes qui n’ont pas de salaire suffisant pour souscrire à une retraite privée et ne peuvent donc pas bénéficier pleinement de leurs années de cotisation dans notre pays. La principale difficulté est la mauvaise interprétation du système de retraite français par l’administration néo-zélandaise. En considérant la pension française comme une retraite d’État, elle la juge comparable à la pension néo-zélandaise. Or la spécificité d’un système contributif comme le nôtre est que la pension reçue est le fruit des années de cotisation des pensionnés. Il serait donc utile

une convention bilatérale de sécurité sociale pourrait permettre de corriger cette situation. Je vous demande de lancer une initiative auprès de nos homologues pour la mise en place d’un accord de sécurité sociale permettant le cumul des pensions de retraite entre nos deux pays. Plus largement, en raison des problématiques spécifiques rencontrées par nos compatriotes établis hors de France, lors du débat

plus de 80 % de la population française expatriée. La décision d’entamer les négociations en vue de signer une nouvelle convention repose sur une analyse d’impact des flux de population entre les pays concernés, mais aussi de compatibilité entre notre régime de sécurité sociale et celui de notre potentiel partenaire. Il convient aussi d’en évaluer l’équilibre financier. En l’absence d’un accord de coordination des systèmes de sécurité sociale et en application des articles 762-1 à L. 762-10 du code de la sécurité sociale, les Français résidant à l’étranger ont la possibilité de bénéficier de prestations du régime de sécurité sociale française en cotisant à la Caisse des Français de l’étranger, notamment pour le risque vieillesse. Selon les derniers recensements, environ 5 000 Français sont inscrits auprès du consulat. De son côté, la communauté néo-zélandaise en France est estimée à 1 400 personnes. La Nouvelle-Zélande n’a pas sollicité des autorités françaises l’ouverture de négociations dans le domaine de la sécurité sociale. Cela n’a donc pas été envisagé à ce stade. C’est pourquoi la question du cumul d’une retraite française et du n’a pas encore fait l’objet d’une analyse par les autorités françaises compétentes. Dans un premier temps, il est nécessaire de mieux expliquer aux autorités néo-zélandaises la nature des pensions de retraite françaises, qui, comme vous l’avez rappelé, sont le résultat des cotisations versées par le bénéficiaire et non une aide attribuée par l’État,

de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 (texte de